avis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

biodiversité » ? Le programme 362 allouait déjà des crédits à la rénovation des bâtiments publics, au développement du tri et à la valorisation des déchets, à la densification et au renouvellement urbain- c'est le fond Friches -, à la restructuration des locaux d'activité,

les programmes budgétaires relatifs aux transports affichent une forme de continuité pour l'année 2023. Cela pourrait sembler rassurant dans la mesure où les investissements dans les infrastructures de transport sont, par nature, des opérations pluriannuelles, qui exigent constance et permanence. Pourtant, cette situation nous inquiète. Elle nous inquiète, car nous savons à quel point les besoins d'investissements dans les infrastructures de transport sont criants, à quel point ces infrastructures sont dégradées et à quel point il faudrait plus de moyens. Nous sommes d'autant plus préoccupés que cette situation tend à s'aggraver ; le réseau ferroviaire en est le meilleur, ou plutôt le pire des exemples. Le Gouvernement avait annoncé un signe sur les infrastructures ferroviaires, mais nous avons eu beau chercher, nous n'avons rien trouvé. Pis, le ministre chargé des transports a annoncé comme objectif le maintien du niveau actuel du réseau ferroviaire. Un tel objectif nous paraît particulièrement peu ambitieux quand on connaît l'état de dégradation du réseau. À cet égard, je rappelle que l'âge moyen du réseau en France est de 30 ans, contre 17 ans en Allemagne. Cet objectif se révèle de surcroît improbable en raison des effets de l'inflation, dont nous reparlerons. Le Gouvernement nous renvoie à l'année prochaine, dans l'attente des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures (COI), qui devront conduire à une nouvelle programmation de financement présentée au Parlement d'ici à la mi-2023, comme l'impose la loi d'orientation des mobilités (LOM). Sans présumer la conclusion de ses travaux, on sait déjà qu'ils impliqueront un véritable exercice de confrontation à la réalité : celle d'un mur d'investissements colossal. À cet égard, il est déjà clair que l'enveloppe qui avait été prévue dans la LOM pour la période 2023-2027 sera nettement insuffisante, si on ajoute les projets de RER annoncés par le Président de la République, dont nous reparlerons plus tard. Enfin, cette continuité apparente nous préoccupe d'autant plus dans la période actuelle d'inflation, où les coûts des chantiers explosent. Le maintien des trajectoires de financement en euros courants serait une catastrophe pour la régénération du réseau ferroviaire. Alors que les investissements sont déjà notoirement insuffisants, comme je l'ai indiqué, les conséquences de l'inflation pourraient s'élever à 500 millions d'euros en année pleine.

S'il n'est pas révisé, notre réseau ferroviaire pourrait se déliter et les ralentissements récurrents que l'on observe jusqu'à présent sur les petites lignes pourraient se diffuser sur les lignes les plus circulées. Face à ce constat, nous avons acquis la conviction qu'il n'est pas raisonnable d'attendre l'année prochaine. C'est pour cette raison que nous défendons, au nom de la commission des finances, un amendement visant à augmenter dès cette année les investissements de SNCF Réseau dans les infrastructures ferroviaires.

Nous sommes d'ailleurs scandalisés par l'attitude des sociétés concessionnaires d'autoroutes, qui, parce qu'elles sont en conflit avec l'État concernant la taxe d'aménagement du territoire, refusent toujours de verser, pour la deuxième année consécutive, la contribution de 60 millions d'euros qu'elles C'est proprement scandaleux ! Par ailleurs, lors de nos auditions, nous avons été très surpris d'apprendre que, cette année, l'Afit France a été limitée non par ses recettes, mais par sa capacité à dépenser les crédits qui lui sont alloués. Cette situation est tout à fait ubuesque au regard des besoins d'investissements dans les infrastructures de transports. Elle s'expliquerait, selon nos interlocuteurs, notamment par le fait que, dans le cadre du plan de relance, de nombreux maîtres d'ouvrage ont présenté des calendriers

En 2023, grâce aux crédits du plan de relance, le montant prévisionnel des dépenses de l'Afit France est certes inédit, puisqu'il atteindra 3,8 milliards d'euros, mais, compte tenu des révisions à la baisse qui interviennent de façon récurrente au fil des budgets rectificatifs,

Le projet de loi de finances pour 2023 maintient les nouvelles aides d'exploitation en faveur du fret ferroviaire. C'est heureux, car, sans ces aides, nous n'atteindrons jamais l'objectif que l'on s'est fixé de doubler la part modale du fret ferroviaire d'ici à 2030. Cependant, les opérateurs de fret sont aujourd'hui menacés par le péril des prix de l'énergie, comme bien d'autres. L'an dernier, une aide exceptionnelle de 26 millions d'euros avait permis de couvrir une part de leurs surcoûts. En 2023, ces surcoûts devraient quadrupler pour atteindre 400 millions d'euros. Cette situation pourrait donc réellement mettre le secteur en péril. Aucune aide n'est prévue dans le PLF, mais nous avons appris que le ministère des transports et le secteur échangent pour concevoir un dispositif, sur lequel nous aimerions obtenir des précisions. Au-delà des aides à l'exploitation, l'enjeu majeur est l'investissement dans les infrastructures, comme l'a rappelé Hervé Maurey. Au total, 10 milliards d'euros seront nécessaires d'ici à 2030, spécifiquement pour le fret. Malheureusement, le contrat de performance de SNCF Réseau est très minimaliste sur ce sujet, ce qui semble admis par tous. En tout cas, cela ne suscite aucune réaction à ce jour. Nous vous avons déjà fait part de notre profonde inquiétude s'agissant de la régénération du réseau ferroviaire. Mais, au-delà de cette régénération, nous ne comprenons pas qu'aucun financement ne soit prévu pour moderniser notre réseau. Nous voulons bien sûr parler des programmes de commande centralisée du réseau et d'ERTMS, le système européen de signalisation ferroviaire, deux innovations qui sont sources de gains de performance considérables, de retours sur investissement et que la plupart de nos voisins européens ont déjà déployées. En plus de l'amendement que mon collègue et moi-même avons déposé visant à abonder en urgence l'enveloppe de régénération du réseau ferroviaire, la commission des finances défend une majoration, bien plus modeste, de 4,6 millions d'euros de la subvention versée à l'Autorité de régulation des transports. Celle-ci s'est vu confier de nouvelles missions et de nouveaux effectifs ces dernières années, sans que l'État lui donne les moyens de les financer, alors que ses réserves s'amenuisent. Cette situation est d'autant moins soutenable

Enfin, nous ne pouvons conclure notre présentation des crédits relatifs aux transports de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » sans manifester notre incompréhension, pour ne pas dire plus, après les dernières déclarations du Président de la République concernant les projets de RER métropolitains.

Les contradictions manifestes entre les déclarations du Gouvernement et cette annonce témoignent non seulement d'un manque de considération pour le Parlement, mais, plus grave encore, elles affectent la crédibilité du message public, dans une confusion généralisée et entretenue.

De notre côté, nous assumons de répondre à l'urgence en faisant un indispensable effort, souvent annoncé par le Gouvernement, mais jamais concrétisé, en faveur des infrastructures ferroviaires gravement menacées par le choc inflationniste. Comme

accroître la transparence des coûts, notamment en abordant enfin la question du poids des péages dans notre pays et celle des tarifs pour développer une politique de l'offre. Bien que nous ayons émis d'importantes réserves sur

de l'information géographique et forestière (IGN) et de Météo-France. Depuis plus de dix ans, ces opérateurs avaient connu des baisses ininterrompues d'effectifs et de moyens financiers.

budgétaire trouve parfois ses limites et j'ai pu constater, à l'occasion des deux derniers contrôles budgétaires que j'ai effectués au nom de la commission des finances, que ces limites avaient été atteintes pour Météo-France et qu'il était nécessaire de donner un peu d'air à l'IGN.

Pour Météo-France, c'était d'autant plus nécessaire que cet opérateur est sans doute le plus affecté par la hausse du coût de l'énergie : ses supercalculateurs sont très gourmands en électricité.

Celui-ci porte des enjeux majeurs en matière de souveraineté des données géolocalisées. Cet établissement devait se transformer pour ne pas être marginalisé ou risquer de disparaître. La trajectoire

Le modèle économique de l'IGN, qui repose sur l'obtention de grands contrats d'accompagnement des politiques publiques, n'est pas sans risque. Il nous faudra en évaluer la viabilité, notamment à l'horizon 2025.

Ses ressources provenant non pas du budget de l'État, mais du secteur du transport aérien, qui paie des redevances pour l'utilisation de ses services, chacun comprend que l'équilibre budgétaire a été quelque peu malmené ces dernières années en raison de la baisse du trafic.

le secteur est convalescent, il se trouve désormais exposé à la crise du prix de l'énergie. La compétitivité des compagnies reste fragile. Ce paramètre, trop souvent éludé, doit être pris en compte dans l'équation globale.

pour 2023 intervient dans un contexte de crise énergétique inédit. Notre commission approuve, sur le principe, la prolongation du bouclier tarifaire, la baisse de la fiscalité énergétique et la revalorisation des crédits alloués à la rénovation énergétique, à la mobilité propre ou à certains opérateurs de l'État, dont l'Ademe et l'Agence Satisfaits de la reprise de nos recommandations passées, nous appelons à concrétiser ces annonces. Pour autant, notre commission relève que la hausse des crédits du programme 174, « Énergie, climat et après-mines », est due à un effet de périmètre et que la baisse de ceux du programme 345, « Service public de l'énergie à la flambée des prix. De plus, nous nous inquiétons de l'application des volets énergie des plans France Relance et France 2030 : pour 2023, les engagements de crédits n'atteignent pas 15 % de ceux qui sont prévus pour le premier, 25 % pour le second.

Notre commission déplore également plusieurs angles morts des crédits : ainsi, la revitalisation des territoires touchés par les arrêts de centrales n'est plus soutenue ; de plus, les dispositions budgétaires et fiscales ne sont pas assez favorables au nucléaire, à l'hydroélectricité, à l'hydrogène, au biogaz et aux biocarburants. Dans ce contexte, le Sénat a adopté voilà quelques jours plusieurs amendements fiscaux, que j'ai présentés à titre personnel. Ils ont permis d'abaisser la fiscalité sur le biogaz et l'électromobilité, mais également de revenir sur un article du Gouvernement

Compte tenu de la gravité de la crise énergétique, notre commission a adopté six amendements budgétaires visant à garantir l'éligibilité des collectivités territoriales et des TPE-PME à l'amortisseur électricité ; à augmenter de 800 000 euros les moyens de la CRE pour contrôler le bouclier tarifaire ; à prolonger l'éligibilité des ménages intermédiaires à MaPrimeRénov' ; à relever de 120 millions d'euros les crédits

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis de sagesse sur les crédits relatifs aux transports ferroviaires, fluviaux et maritimes pour l'année 2023.

Face à votre réalité politique, qui canalise la contre-performance ferroviaire, nous souhaitons faire du train le pilier de la mobilité pour enfin vitaminer le report modal. Faute de moyens supplémentaires, la réalité hypothétique des « RER Macron » est une « remontada » de façade, rangée pour l'instant à quai de gare.

S'il faut améliorer les déplacements métropolitains, il faut également répondre aux besoins de la France périphérique. Dans ce cadre, nous avons défendu ici la baisse de la TVA à 5,5 %, en guise d'amortisseur, autant pour les autorités organisatrices de la mobilité que pour les usagers. Il s'agit, enfin, d'appliquer ce que le Sénat a inscrit dans la loi, le doublement de la part du fret ferroviaire et fluvial, et de rendre plus compétitives et vertueuses nos infrastructures portuaires. Ce projet de budget permet-il de faire face à ces difficultés ? Nous sommes encore loin du compte. Les collectivités prennent largement leur part. À l'État, dans sa stratégie de souveraineté, de tracer le chemin.

Aussi, je défendrai une enveloppe de 150 millions supplémentaires en faveur de l'investissement ferroviaire, même si je suis bien conscient qu'il en faudrait bien plus. Nous souhaitons également doper les capacités sous-exploitées du transport fluvial, qui a démontré sa résilience.

Agir sur les mobilités, c'est conjuguer aménagement du territoire et réponse aux défis sociétaux. Plus on propose une diversité de solutions, mieux on répond à nos exigences de services publics. Telle est l'ambition portée par notre commission.

la clé de l'équilibre de ce budget annexe, ce sont des recettes gouvernées par le niveau du trafic aérien, qui dépend lui-même du prix des billets d'avion et de la psychologie des voyageurs.

des installations de contrôle aérien ne risque-t-elle pas de remettre en cause le rééquilibrage prévu, comme c'est le cas pour de nombreuses entreprises et collectivités ? Deuxièmement, la France est l'un des deux leaders mondiaux de la construction aéronautique et peut décarboner 50 % de la flotte mondiale. Nous sommes également pionniers dans la réglementation environnementale, face à ses effets et avec les nouveaux mandats d'incorporation des kérosènes durables au niveau national ou européen. Notre talon d'Achille, c'est notre retard pour produire et distribuer ces biocarburants,

zéro émission pour les opérations au sol et production d'hydrogène vert, gazeux pour les engins au sol et liquide pour les futurs avions, qui seront opérationnels en 2035. Enfin, les 8 à 9 millions de riverains des aéroports, eux aussi, travaillent plus qu'avant à domicile. Les nuisances perçues peuvent donc parfois augmenter même quand le trafic diminue. Nous approuvons les nouvelles trajectoires plus économes en carburant, mais les descentes continues impliquent de voler plus longtemps à basse altitude. Le financement des travaux d'isolation, qui est assis sur une taxe indexée sur le trafic, n'avait pas prévu ces évolutions, et les pertes de recettes se sont accumulées. Une nouvelle rallonge budgétaire est donc souhaitable, d'autant que le bon sens plaide pour le couplage de l'isolation acoustique et thermique, à double efficacité environnementale.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable sur l'adoption des crédits relatifs aux transports routiers de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », sous réserve de l'adoption de treize amendements.

j'aborderai la question majeure de la décarbonation du parc de véhicules. Le déploiement, à court terme, des zones à faibles émissions mobilité, conjugué à la définition d'objectifs ambitieux de fin de vente des véhicules thermiques à l'échelle nationale et européenne, impose de mieux soutenir les ménages,

de louer des véhicules électriques. En effet, à ce stade, celui-ci ressemble davantage à une coquille vide qu'à une véritable solution d'accompagnement pour nos concitoyens. Monsieur le ministre, vous demandez aujourd'hui au Parlement de se prononcer sur un dispositif mobilisant des montants substantiels,

pour l'acquisition de véhicules moins polluants, et cela sans qu'il soit besoin d'inventer de toutes pièces de nouveaux dispositifs. Mon deuxième point d'alerte concerne l'état de nos infrastructures routières. Je pense non seulement aux voies, mais également aux ouvrages d'art.

les ouvrages d'art, ne nous arrêtons pas aux constats du programme national Ponts, qui a certes permis une réelle avancée, mais qui doit se poursuivre par des travaux de réparation des ouvrages les plus dégradés.

vise surtout à absorber la hausse tendancielle des dépenses contraintes de ce programme, au sein duquel les subventions pour charges de service public distribuées à différents opérateurs, comme l'Ademe, l'Anses représentent les deux tiers des crédits, en progression de 5 % par rapport à 2022. Je note avec satisfaction que les baisses d'effectifs au sein du pôle ministériel de la transition écologique marquent une pause, après une décennie de diminution continue. Sur ce sujet, je ne puis que regretter de nouveau le manque de précision concernant les effectifs des inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Chaque fois que je pose la question, j'obtiens une réponse différente ! Ce n'est pas très rassurant ... Il semble Il semble également y avoir un problème structurel de vacances de postes. Je souhaite, monsieur le ministre, que le Gouvernement travaille sur ce sujet, car il s'agit de services essentiels pour assurer la conciliation des objectifs de développement industriel et de protection de l'environnement et de la santé des populations. En outre, sans un travail sur l'attractivité des postes, le Gouvernement ne pourra pas honorer sa promesse, faite à la suite de l'incendie majeur des usines Lubrizol et Normandie Logistique en 2019, de renforcer l'inspection des ICPE, alors que les enjeux sont extrêmement

entend marquer l'importance de la prévention du risque d'inondation, auquel 17 millions de nos concitoyens et 40 % de nos emplois sont exposés,

avis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour présenter en trois minutes mon avis budgétaire, j'axerai mon intervention sur la question fondamentale de l'eau. En effet, la sévérité des épisodes caniculaires a démontré, s'il en était encore besoin, la centralité de la question de la ressource en eau dans notre pays. Le programme 113 est le support de financement budgétaire de la politique de l'eau : 21 millions d'euros de crédits de paiement lui sont consacrés pour 2023, avec notamment 900 000 euros pour la mise en oeuvre des préconisations du Varenne agricole de l'eau. La modicité de ce montant m'interpelle, au regard des défis posés par l'adaptation de notre modèle agricole à la nouvelle donne climatique. Un autre point de vigilance, déjà mis en avant sur de nombreuses travées de notre assemblée, porte sur la question des ressources affectées aux agences de l'eau, avec le fameux plafond mordant, c'est-à-dire l'écrêtement des ressources affectées aux agences au-delà de 2,2 millions d'euros et le versement de l'excédent au budget général. Ce mécanisme est à l'origine de plusieurs effets pervers : le taux des taxes est modulé pour s'ajuster à ce plafond, faussant ainsi le signal-prix du coût de l'eau facturé aux usagers et suscitant une tarification qui n'incite pas forcément à la sobriété des usages.

La vétusté croissante des réseaux est à l'origine d'un taux de fuite estimé à 20 %, soit 1 milliard de mètres cubes par an, ce qui est considérable. Elle s'explique par un sous-investissement chronique, récemment évalué à 4,6 milliards d'euros par an. Je note que 50 millions d'euros de crédits supplémentaires ont été consacrés à la rénovation des réseaux d'adduction dans le second projet de loi de finances rectificative pour 2022. C'est un signal positif, mais les montants ne sont toujours pas à la hauteur des défis. Il est dès à présent nécessaire d'accroître la résilience hydrique de notre pays, dans un contexte climatique incertain. Je regrette donc que cette priorité ne ressorte pas plus clairement de l'analyse des crédits de la mission qui nous occupe,

À la veille de la COP15 consacrée à la biodiversité, cet écart entre les ambitions affichées et les moyens budgétaires alloués mérite d'être pointé. Les aires protégées sont un bel outil de protection de la biodiversité et un levier de l'attractivité de nos territoires. Elles méritent d'être financées à la hauteur des bénéfices qu'elles suscitent, comme des services qui y sont rendus par la nature. Il est important que la France mette en cohérence ses discours internationaux et ses actions sur le terrain national. Nation verte, elle se doit d'être exemplaire. Nous serons vigilants et nous comptons sur vous, monsieur le ministre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous présenterai succinctement l'avis exprimé par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » relatifs au développement des énergies renouvelables et à la rénovation énergétique des bâtiments. Je commencerai par les énergies renouvelables. À cet égard, la France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint l'objectif fixé pour 2020. Le déploiement des énergies renouvelables est pourtant doublement nécessaire à notre pays, d'une part, atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et, d'autre part, pour préserver notre sécurité d'approvisionnement. Ce retard est également dommageable d'un point de vue financier. Fait exceptionnel dans un contexte budgétaire tendu, le développement des énergies renouvelables

du prix de l'électricité et du gaz. Ce sont ainsi 39,4 milliards d'euros qui entreront dans les caisses de l'État pour l'exercice budgétaire à venir ! La situation est bien différente pour la chaleur renouvelable, qui nécessite aujourd'hui un soutien public accru. Je vous proposerai donc, au nom de notre commission, un amendement tendant à porter le montant du fonds Chaleur de 520 milliers d'euros à 700 millions d'euros, ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de de l'énergie. J'en viens au second thème de cet avis, à savoir la rénovation énergétique des bâtiments. Si le PLF pour 2023 consacre une pérennisation bienvenue de MaPrimeRénov', notre commission déplore le bilan énergétique insuffisant de ce dispositif. Nous avons calculé que les économies d'énergie permises par MaPrimeRénov'ne représenteraient, en 2021, que 0,15 % de la consommation totale du parc résidentiel. À ce rythme-là, nous en avons pour des décennies ! La commission estime donc nécessaire d'orienter plus massivement les aides vers les rénovations globales ou multigestes, à moyens constants. Le déploiement du service France Rénov'et, à partir de 2023, d'un réseau d'accompagnateurs agréés doit également soutenir des travaux ambitieux. La massification de la rénovation énergétique passera parallèlement par la structuration des filières de rénovation et la montée en compétences des professionnels. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, les réserves de la commission portent plus sur l'exécution que sur les montants retenus par le PLF. Elle a donc émis un avis favorable sur l'adoption des crédits relatifs à la transition énergétique et climatique,

relatif au fonds Chaleur. Très bien ! Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de quinze minutes pour intervenir.

Que faisons-nous du reste du territoire ? Que faisons-nous de la ruralité ? Que faisons-nous de ces 22 millions de Français qui n'ont d'autre solution que d'avoir une, voire deux voitures par ménage et qui subissent par conséquent l'inflation, avec un gazole à plus de 2 euros le litre ?

Fort heureusement, concernant le défi écologique, nous n'en sommes plus à l'étape de la prise de conscience. Malheureusement, cela signifie aussi que le dérèglement climatique est visible. Cette année, nous l'avons subi de plein fouet et sur l'ensemble du territoire. Le gel a tout d'abord attaqué le vignoble. La canicule, ensuite, a endommagé nos cultures et fait souffrir nos élevages. Depuis lors, la sécheresse a sévi- c'est d'ailleurs toujours le cas dans quelques territoires -, et certaines de ses conséquences sont désastreuses. Alors que nous nous pensions épargnés, nous avons dû faire face à de violents incendies de forêt au nord même de la Loire. Le Maine-et-Loire, qui nous tient à coeur particulièrement, monsieur le ministre, a été cet été l'un des départements les plus touchés. Au total, plus de 2 500 hectares sont partis en fumée en l'espace de quelques semaines. À Baugé-en-Anjou, 1 500 hectares ont brûlé en seulement trois jours. Je salue et remercie tous nos pompiers qui ont affronté ces feux, partout en France, ainsi que nos concitoyens, particulièrement nos agriculteurs, qui ont également apporté une aide précieuse. Notre groupe prend sa part de cet effort, en travaillant sur des mécanismes concrets, à l'image de l'agrivoltaïsme ou de nos propositions sur la forêt. En tant qu'élus nationaux ou locaux, nous avons chacun notre rôle à jouer. Continuer à nous alerter et à nous former sur les enjeux de la transition écologique est nécessaire. Mettre à disposition des élus un outil pour cela, afin qu'ils s'en emparent, va incontestablement dans le bon sens. D'ailleurs, le fonds vert, qui leur donne des moyens d'action adaptés à leur territoire, procède de cet état d'esprit. Nous ne pouvons que saluer cette initiative, dans la chambre des territoires Aux bouleversements climatiques se sont ajoutées la guerre en Ukraine et les conséquences énergétiques que nous endurons. Le groupe Les Indépendants salue les réponses conjoncturelles, qui ont été décrites par les très nombreux rapporteurs spéciaux et pour avis,

L'énergie est cruciale pour notre compétitivité. Notre tissu industriel, notre agriculture et, plus généralement, nos modes de vie en sont dépendants, nous le voyons bien à l'approche de l'hiver.

Cette mission montre tout le chemin qu'il reste à parcourir dans ce domaine. Il nous faut travailler massivement sur nos infrastructures. Les modes de mobilité sont très variés selon les territoires. Notre réseau ferré doit rester performant et vecteur de transition. Nos voitures, si nécessaires à des millions de Français dans nos territoires, doivent devenir plus propres. Le travail dans ce domaine est immense. Il faut agir bien, et pour longtemps. Tous les programmes de cette mission tendent vers la même conclusion : nous allons devoir nous adapter, et il faut nous en donner les moyens. Pour décarboner, il va falloir innover et trouver des solutions disruptives. Nous devrons être acteurs de prévention, tout en réduisant les problèmes auxquels nous faisons déjà face. Pour cela, il faut investir. À cet égard, je salue à la fois la hausse significative des crédits de la mission et la stabilité dans les effectifs, qui augmentent même dans certains secteurs. La transition est, en quelque sorte, une révolution. Elle est nécessaire. Nous devons donc impérativement la rendre possible et acceptable pour tous. Il faut voir loin pour faire bien, si j'ose dire. Monsieur le ministre, la feuille de route est belle, mais elle n'est pas sans obstacle. Il faut inventer à nouveau nos modes de vie. Vous l'aurez compris, le groupe Les Indépendants - République et Territoires votera les crédits de cette mission.

Il nous faut donc envisager la pertinence du budget de la mission « Écologie développement et mobilité durables » à l'aune de son adéquation à ces défis. Parmi les nouveautés de l'année figure le fameux fond vert pour les collectivités territoriales, porté à 2 milliards d'euros par l'Assemblée nationale.

vous connaissez aussi, monsieur le ministre, les inquiétudes des élus locaux sur les difficultés de fonctionnement de leurs collectivités territoriales, notamment, mais pas seulement, du fait de la flambée des coûts de l'énergie, qui remet en cause leur capacité d'investissement.

Surtout, le montage des dossiers butera, comme d'habitude, sur les difficultés d'ingénierie et d'animation territoriale, qui sont pourtant le coeur d'une transition territoriale réussie. Pour faire face à cet enjeu, nous avons de nouveau adopté à la quasi-unanimité, ici au Sénat, une dotation de fonctionnement climat, en première partie du présent projet de loi de finances.

mais récupérables sur le long terme, notamment par les économies réalisées sur l'efficacité énergétique. Il faudrait même certainement prévoir une comptabilité spécifique pour éviter de stigmatiser cet endettement nécessaire l'ombre de Bercy plane et menace toujours l'effort de transition nécessaire des territoires. En ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments, les dispositifs d'aide ne sont pas opérationnels aujourd'hui, tout le monde

Pour le ferroviaire- mon collègue Jacques Fernique y reviendra -, malgré la reprise de 35 milliards d'euros de dette de SNCF Réseau et les fonds de relance vers le fret et les trains de nuit, il manque encore au moins 1 milliard d'euros par an. Le contrat de performance 2021-2030 établi entre l'État et SNCF Réseau a fait beaucoup de déçus. Concernant enfin le ministère lui-même, on peut se féliciter

d'effectifs et de baisse de budgets cumulés. Le dernier rapport d'I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat, est on ne peut plus explicite sur le sujet : entre 2014 et 2021, le Cerema a perdu 633 emplois, Météo-France 602 et l'IGN 254 ! Ces réductions ont été tellement importantes qu'il sera impossible de reconstituer ces emplois à court terme. Or le manque d'accompagnement au sein de l'État en matière environnementale et de transition écologique se fait déjà largement ressentir. Le temps me manque, mais j'aurai aussi un mot pour les agences de l'eau : il faut aller au-delà de la sanctuarisation de leur budget. Le rehaussement du plafond mordant est une piste intéressante, mais encore insuffisante. Nous devons augmenter et pérenniser les moyens dont elles disposent pour leur pour leur action en faveur du grand cycle de l'eau et de la biodiversité. Il nous faut certainement une fiscalité dédiée renforcée en matière de protection de la biodiversité. La stratégie nationale pour les aires protégées n'a pas encore trouvé de financement à la hauteur des objectifs, et nous sommes encore très loin du compte pour les zones de protection forte. mes chers collègues, nous aurions préféré acter un tournant budgétaire décisif dans la politique gouvernementale en faveur de l'écologie. Aussi les amendements proposés par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires n'ont-ils finalement qu'un but : mettre la loi et les financements des politiques publiques en cohérence avec les engagements pris par la France. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette année, comme la précédente, a mis en lumière que le dérèglement climatique est, pour celles et ceux qui en douteraient encore, encore, une réalité tangible, illustrée par une série de canicules, des feux de forêt gigantesques, des sécheresses record et des épisodes pluvio-orageux violents à répétition. Par ailleurs, la guerre en Ukraine et l'aggravation de la crise énergétique qui en résulte ont entraîné des difficultés sociales et économiques pour une écrasante majorité de nos compatriotes, confrontés à une nette augmentation des prix de l'énergie et du carburant. Ces enjeux nous obligent : loin de sombrer dans le fatalisme et la résignation, notre pays doit conduire une politique écologique et environnementale volontariste aux échelles nationale, européenne et mondiale. Ces enjeux et ces difficultés nouvelles nous rappellent combien il est essentiel de placer notre pays sur la trajectoire de la neutralité carbone à l'horizon 2050 et de le sortir de sa dépendance aux énergies fossiles. Ces enjeux, ce sont ceux de la mission que nous examinons aujourd'hui, présentés au travers des différents programmes portant les moyens financiers historiquement élevés que l'État a souhaité consacrer dans le PLF pour 2023 et dans la trajectoire pluriannuelle, ici présentée jusqu'en 2025. Pour parvenir à ces objectifs ambitieux, mais impératifs, la transition écologique et énergétique doit être accélérée, avec une évolution des politiques portées par l'État, au travers tant des missions directement impulsées par les ministères de la transition écologique et de la transition énergétique que de celles des autres administrations publiques. Cette démarche stratégique nationale et interministérielle doit permettre d'améliorer la résilience de nos écosystèmes, de renforcer la sobriété de nos modes de vie, de préserver la biodiversité et les ressources primaires, de conduire une transition socialement juste et de développer les filières vertes sur les territoires. Oui, la reterritorialisation de la transition écologique est non pas un luxe, mais une nécessité ! Je veux, à ce stade, mettre l'accent sur le fonds pour l'accélération de la transition écologique dans les territoires, qui répond à la succession des crises climatiques. Ce fonds doté de 2 milliards Ce fonds doté de 2 milliards d'euros, soit 500 millions d'euros supplémentaires, permettra de soutenir les collectivités territoriales et leurs opérateurs dans leurs investissements, leurs aménagements, leurs choix d'urbanisme et les multiples services qu'ils proposent. Il portera de manière déconcentrée le financement du déploiement de la stratégie nationale pour la biodiversité dans les territoires. Affronter la hausse des coûts de l'énergie, c'est accélérer la sortie des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables. Nos débats récents ont prouvé que nous pouvions converger sur le sujet. Cette préoccupation de transition écologique, énergétique et solidaire, on la retrouve au coeur de la politique maritime de la France- deuxième puissance mondiale dans ce domaine, je le rappelle -, portée par le programme 205 dédié au développement durable des activités maritimes, au plus près des usagers de la mer et des territoires fluviaux, ainsi qu'au développement de nos ports maritimes, afin de limiter le transit routier. Toutefois, nous le savons, lutter contre notre dépendance aux énergies fossiles passe par une nouvelle façon de se déplacer. Tel est l'objet du programme 203, dont 90 % des crédits soutiennent le développement de mobilités décarbonées : le ferroviaire, mais aussi le fluvial, le portuaire, le transport combiné et les mobilités douces. Au passage, la trajectoire d'investissements prévue par la loi d'orientation des mobilités pour la période 2019-2023 a été respectée, et même dépassée. Ce fait mérite d'être souligné. de transport (Afit France) pour 2023 porte le budget global dédié aux transports terrestres et fluviaux à plus de 9,3 milliards d'euros, en augmentation de 6 %. Les engagements pour le secteur ferroviaire sont notables, même si l'effort de rattrapage reste pour partie devant nous après des décennies de sous-investissement. Le transport ferroviaire et le fret sont deux thématiques sur lesquelles le Gouvernement s'est fortement engagé durant la législature précédente, et je ne doute pas qu'il continuera à le faire, si j'en juge par ses annonces récentes. S'agissant du transport fluvial, le PLF traduit un effort soutenu, grâce au plan de relance, à hauteur de 175 millions d'euros. Le contrat d'objectifs et de performance signé au printemps 2021 entre Voies navigables de France (VNF) et l'État a fixé une trajectoire ambitieuse d'investissements en régénération et modernisation du réseau fluvial. Ces actions, auxquelles n'étaient consacrés en moyenne que 150 millions d'euros par an avant 2021, ont bénéficié de 230 millions d'euros en 2021 et 2022. Ce niveau sera maintenu en 2023, et la trajectoire ambitieuse s'accélérera à partir de 2026 et 2027. Quant au transport aérien, il sort d'une crise sans précédent liée à l'épidémie de la covid-19. Le trafic aérien français a chuté de 70 % en 2020 et de 61 % en 2021 par rapport à 2019. En août dernier, il a retrouvé 90 % de son niveau enregistré en août 2019. Les mesures de soutien public mises en place par le Gouvernement dès le début de la crise sanitaire ont été indispensables à la survie du secteur. Pourtant, la régulation du transport aérien joue un rôle essentiel dans la décarbonation. Beaucoup de travail reste à faire ; il nous faut continuer à progresser dans l'offre de solutions alternatives à l'avion, dans les efforts de décarbonation du secteur, dans la sensibilisation des consommateurs le développement du ferroviaire- ce week-end, je dois avouer que c'est un peu compliqué ... Ce défi de la transition écologique, nous avons à le relever ensemble. Nous ne le relèverons pas les uns contre les autres, ni les uns au détriment des autres. Chacun est dans ses responsabilités, chacun est dans son rôle, même si, en quelque sorte,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du projet de loi de finances intervient dans un contexte particulier, celui d'une France en feu et d'une Europe en guerre. Incendies, températures record, alertes sécheresse- y compris dans mon département du Nord, c'est pour dire ! -, nappes phréatiques asséchées, manque d'eau c'est aussi la guerre en Ukraine, qui met en lumière notre dépendance à l'égard de puissances étrangères et des énergies fossiles. Ce moment si particulier devrait nous amener à répondre aux enjeux de ce que l'on peut appeler le défi,

Au pied du mur, face au risque de pénurie, le Gouvernement n'a trouvé comme réponse que des retours en arrière. Avec le projet de loi relatif à l'accélération de la production des énergies renouvelables, c'est le terminal méthanier du Havre, le gaz de schiste et les centrales à charbon qui ont fait leur triste retour. Nous déplorons grandement le manque d'anticipation et de vision d'ensemble du Gouvernement pour que la France se dote d'une réelle politique environnementale. L'examen de cette mission dite « Écologie » le confirme : le virage tant attendu et tant annoncé n'aura pas lieu. Si le budget est en hausse, c'est bien parce qu'il y a financement de mesures d'urgence liée à la crise énergétique bouclier tarifaire et soutien aux effacements de consommation énergétique. Mais le budget ne comporte aucune réforme structurelle permettant de financer l'accélération de la transition écologique. Ainsi, on constate que les crédits alloués au transport routier, notamment à l'entretien des routes, sont en forte hausse, alors que les crédits dédiés aux transports collectifs et combinés sont en baisse.

Les perturbations en chaîne se multiplient, de nombreux usagers partout dans les territoires, notamment dans les Hauts-de-France, souffrent quotidiennement de désagréments. La rénovation des voies ferrées, âgées de 30 ans en moyenne en France, devient de plus en plus urgente.

de ce qui est nécessaire au regard des enjeux qui seront largement évoqués lors de la COP15 biodiversité à Montréal. Surtout, alors que la France entend incarner un leadership fort dans ce combat, quelle crédibilité accorder à notre parole quand ces financements restent notoirement insuffisants Enfin, j'aurai un mot particulier pour le nouveau programme « fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires », ou fonds vert il va dans le bon sens, car le rôle des collectivités est effectivement fondamental dans cette transition écologique, mais nous restons encore dans l'attente de précisions sur la manière dont il sera

de prendre en compte l'accélération alarmante du réchauffement climatique. Néanmoins, une fois encore, il est difficile de considérer que la COP27 fut un succès. Comme le dit très justement Jean-Marc Jancovici, une COP, c'est énormément de discussions pour finir par arriver à un texte qui est souvent malheureusement une déclaration d'intention. Le nombre des lobbyistes des énergies fossiles à la COP27 dépasse d'ailleurs le total des représentants des dix pays les plus touchés par le changement climatique. Avec presque 32 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 30,5 milliards d'euros en crédits de paiement, le budget en faveur de l'écologie affiche certes une hausse notoire, mais intègre près de 9 milliards d'euros destinés à financer des aides aux consommateurs, notamment le bouclier tarifaire. il faut le dire, TotalEnergies enregistre des bénéfices record, sans parler des plus de 2 milliards d'euros de dividendes exceptionnels annoncés. Certes, la France a le mérite de se fixer des objectifs ambitieux dans sa stratégie nationale bas-carbone pour contenir les émissions de gaz à effet de serre et la hausse des températures à 2 degrés d'ici à 2050.

ce qui se traduirait par un taux de subvention égal à 25 % ... Dans ces conditions, il est à craindre que ce fonds bénéficie aux collectivités les mieux dotées, à la fois en moyens humains, pour répondre à des appels à projets toujours plus complexes, et en capacité d'investir sur leurs fonds propres, pour répondre à des critères qui, pour le moment, restent assez flous. Le Gouvernement a raison de dire qu'il n'y a pas d'argent magique. Mais l'urgence climatique est là, et bien là. L'été 2022 restera dans les mémoires comme l'été de la fin de l'insouciance. Dans mon département, comme dans d'autres d'ailleurs, au-delà des incendies à répétition, la tempête de grêle incroyablement dévastatrice a provoqué des pertes considérables pour nos agriculteurs et nos concitoyens, dont les maisons sont encore à ce jour habillées de bâches dans le Ribéracois. L'indispensable transition écologique nous oblige à des investissements importants importants et à une plus juste répartition des richesses produites. Avec seulement deux réformes, la suppression de l'ISF et le prélèvement sur les APL, le Gouvernement a pris 1,3 milliard d'euros aux bénéficiaires de l'aide au logement et en a redistribué presque trois fois plus aux plus riches des Français. Contrairement à d'autres pays voisins, la France a refusé de taxer les profits exceptionnels suscités grâce et à cause de la crise. Monsieur le ministre, on ne peut pas parler de transition écologique si l'on ne parle pas de justice sociale ! Nous avons besoin de réformes structurelles : adaptation de nos forêts, de nos bâtiments et de nos infrastructures, rénovation rénovation efficace de nos logements, investissements dans le transport responsable de 30 % de nos gaz à effet de serre ... Tout cela nécessite des investissements importants. Or, dans ce budget, pas de hausse significative des crédits en faveur du ferroviaire, alors que, pour atteindre l'objectif fixé par la stratégie nationale bas-carbone, près de 3 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an seraient nécessaires

La politique de rénovation thermique n'est pas non plus suffisamment ambitieuse, me semble-t-il. Bien qu'il soit abondé dans ce budget, le dispositif MaPrimeRénov'reste insuffisant, dans la mesure où aucun gain de consommation énergétique minimal n'est requis. L'an dernier, seuls 2 500 logements sont sortis du statut de passoires thermiques. Sur plus de 700 000 000 primes accordées en 2021, pour un montant de 2,8 milliards d'euros, seuls 60 000 logements ont fait l'objet d'une rénovation globale. Le reste à charge conduit en effet les ménages à y renoncer. Enfin, cette mission nous est présentée après des échanges riches sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production des énergies renouvelables, adopté en première lecture au Sénat. Or ce projet de loi de finances ne prévoit aucune ligne budgétaire de soutien à ces énergies, qui restent dans le secteur concurrentiel. L'investissement dans les énergies renouvelables reste tributaire du prix de l'énergie, de l'énergie, ouvert à la concurrence. La bifurcation écologique implique une réindustrialisation, des relocalisations et des créations d'emplois. Elle nécessite la reconstruction de filières industrielles françaises dans le renouvelable et la création d'un pôle public de l'énergie, car l'État doit garder la main sur ce que sont nos biens communs au regard des enjeux sociaux, humains, écologiques, de souveraineté et d'indépendance de notre pays. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le groupe CRCE ne votera pas le budget de cette mission.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà parvenus à l'examen d'une mission fondamentale pour l'atteinte de nos ambitions climatiques et environnementales. Les moyens et les crédits portés par les programmes de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » ont en effet vocation à préparer notre pays aux défis immenses de l'adaptation au changement climatique et à atteindre un meilleur niveau de résilience de nos territoires. Par rapport à la loi de finances initiale pour 2022, les autorisations d'engagement de la mission pour 2023 augmentent de plus de 10 milliards d'euros dans le texte transmis au Sénat après l'engagement de l'article 49.3, contre 6,8 milliards d'euros dans le texte initial. Je ne puis que saluer cette amélioration. Parmi les points de satisfaction à noter, ce budget renforce fortement les aides à l'achat de véhicules électriques, ce qui permettra à davantage de nos concitoyens de s'équiper de véhicules propres, dans la continuité des propositions par notre collègue Philippe Tabarot lors des débats sur la loi Climat et résilience. J'appelle néanmoins le Gouvernement à agir au niveau européen, afin de restreindre au maximum ces aides à des véhicules produits en Europe. Il y va de notre souveraineté industrielle. Un point de satisfaction important concerne la stabilité des schémas d'emplois de la mission du pôle ministériel et des opérateurs rattachés ; après une décennie de baisse drastique, il était temps de mettre fin à l'hémorragie Nous savons que la transition écologique sera intensive en moyens humains et nécessitera un pilotage appuyé sur une expertise publique qu'il faut dès à présent conforter, grâce notamment à l'Ademe, au Cerema, à Météo-France ou à l'IGN. Nous serons donc vigilants quant au respect, par le Gouvernement, de sa promesse de préserver les effectifs au cours du quinquennat. Malgré ce budget globalement satisfaisant, il subsiste des points d'inquiétude importants le gigantisme du bouclier tarifaire sur les carburants entraîne un brunissement marqué de la trajectoire environnementale du budget de l'État. Les dépenses défavorables augmenteront de 90 % par rapport à 2022 Je souscris bien entendu au soutien aux ménages modestes face à l'inflation des coûts de l'énergie, mais je déplore l'absence de compensation et les conséquences à moyen terme sur nos efforts de verdissement par ailleurs. La cohérence de nos politiques publiques gagnerait à ce qu'on mette fin à cet « effet Pénélope », qui consiste à défaire la nuit les efforts patiemment accomplis le jour. J'ai un autre sujet de préoccupation important, concernant le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires,

Ainsi, ce fonds vert, qui consiste en réalité davantage en une pérennisation de crédits initialement déployés dans le cadre du plan de relance, comme le fonds Friches, revêt plus d'un effet d'annonce que d'une réelle nouveauté. Par ailleurs, la mise en oeuvre pratique de ce fonds nourrit des inquiétudes concernant le mécanisme d'attribution des aides. À la main des préfets, pour garantir la souplesse de l'attribution des aides, j'aimerais que l'on puisse m'assurer que les communes aux moyens humains limités seront bien en mesure d'y accéder, car ce sont précisément pour celles-ci que les aides présentent l'effet de levier le plus important. Sous le bénéfice de ces observations, je salue la stabilité de ce budget, l'arrêt de l'hémorragie des emplois au sein des opérateurs rattachés, ainsi que la priorité croissante donnée à l'environnement. Je ne saurais trop inviter le Gouvernement à poursuivre dans cette voie. Notre groupe votera en faveur de l'adoption des crédits de cette mission. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après la COP27, l'examen de ce budget nous permet de faire le point sur les principales politiques qui concourent à la réalisation de l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Or on peut légitimement se demander comment les États, de plus en plus endettés, pourront faire face au mur des investissements nécessaires à la transition énergétique et écologique. Cette année constitue donc un tournant sur le plan énergétique. La guerre en Ukraine nous a rappelé notre fragilité et notre dépendance aux énergies fossiles. Cette année, les énergies renouvelables rapportent des recettes à l'État du fait de l'explosion des prix de l'électricité sur les marchés, ce qui nous permet de financer les aides mises en place en France pour répondre à une situation probablement durable blocage des tarifs réglementés, bouclier tarifaire, amortissement électricité, filet de sécurité pour les collectivités territoriales, chèque énergie, etc. Le coût du maintien de l'économie et de la protection contre la précarité et de la paix sociale pour ces quelques mois représente tout de même 45 milliards d'euros, rien que pour le bouclier tarifaire. Mais, on le conçoit parfaitement, on ne pouvait ne rien faire pour préserver les ménages et les entreprises. Après une crise sanitaire ayant paralysé l'économie, celle-ci se trouve néanmoins en perpétuelle perfusion d'argent public. Les collectivités territoriales bénéficieront finalement d'un soutien important au travers des différents dispositifs prévus par les lois de finances initiale et rectificative. Nous y reviendrons plus longuement et plus sereinement lors de l'examen de la proposition de loi qui sera examinée la semaine prochaine. Cependant, l'avenir de ces aides reste flou, alors que les prix de l'énergie ne peuvent que connaître une hausse structurelle. Jusqu'à quand pourra-t-on tenir ce rythme Les mesures adoptées ces derniers mois ne pourront être indéfiniment prolongées. Le Gouvernement a déposé un nouvel amendement visant à rehausser de 6 milliards d'euros les crédits du programme « Service public de l'énergie », dont environ 2 milliards d'euros pour étendre le bouclier tarifaire, y compris rétroactivement, aux structures collectives d'habitat qui avaient été oubliées en 2022. Je me réjouis de cette intégration. Aussi, la responsabilité nous incombe de progresser pour relever le défi historique que nous impose le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité. Il nous faut donc aller vers davantage de sobriété, ce mot que certains n'osaient prononcer et qui, désormais, ne cesse d'être répété. Pour cela, le chantier de la rénovation énergétique des logements et des bâtiments publics et tertiaires devrait constituer une priorité. Le plan de sobriété constitue une première réponse, mais l'ampleur des besoins et la nécessité de développer des compétences et des filières très rapidement ne peuvent que nous donner le vertige. Il aurait fallu dans l'idéal favoriser les travaux lors des mutations des biens ou des changements de locataires. Nous aurions pu voter cette mesure en 2019, lors de l'examen de la loi Énergie-climat, ou encore en 2021, lors de l'examen de la loi Climat et résilience. Pendant ce temps-là, nous continuons à accroître les montants consacrés à MaPrimeRénov'. Certes, cette hausse est bienvenue, mais ces dépenses publiques sont surtout orientées vers des monogestes sans grand effet sur la consommation énergétique des ménages et sur le climat. En matière de transports, si la trajectoire d'investissements de la loi d'orientation des mobilités est en passe d'être respectée, celle qui doit nous conduire vers la neutralité carbone ne l'est pas. La décarbonation de ce secteur repose pour beaucoup sur le développement du transport ferroviaire, qui doit être une solution de rechange à la fois au transport routier et au transport aérien. La compétitivité du secteur ferroviaire repose avant tout sur les investissements qui doivent être consacrés à la régénération et à la modernisation du réseau. Beaucoup reste à faire pour engager le report modal vers le rail. Nous voterons en faveur de l'amendement proposé par la commission visant à allouer 150 millions d'euros supplémentaires à la régénération du réseau. Enfin, je dirai un mot rapide du fonds vert. Au-delà de l'effet d'annonce, nous espérons qu'il ne s'agira pas d'un simple recyclage de crédits précédemment octroyés. Nous aurions souhaité disposer des modalités précises de fonctionnement et d'affectation des crédits avant l'examen du projet de loi de finances. Pour conclure, nous voyons naturellement d'un mauvais oeil les économies proposées par la commission des finances sur cette mission, soit plus de 700 millions On pouvait certes estimer que les actions concernées étaient surdotées, mais ces crédits auraient pu être réaffectés à d'autres programmes visant à financer les transports, les aides à la rénovation énergétique, la préservation de la biodiversité, le renforcement de la prévention des risques ou encore le fonds vert.

sans doute paralyser et scléroser les collectivités locales, quand bien même elles seraient capables de déployer des trésors d'ingéniosité pour résister à cette folie technocratique. Quant aux zones à faibles émissions, le Gouvernement n'en mesure pas toujours le caractère discriminant et excluant pour les habitants du monde rural. Nous avons aussi depuis peu des projets de loi sur la politique énergétique « saucissonnés », comme pour mieux occulter les erreurs majeures commises il y a dix ans concernant les orientations stratégiques de notre pays en matière énergétique- une stratégie de Gribouille qui nous conduira à de probables coupures électriques cet hiver ... Dans le domaine budgétaire, on trouve ici et là les marques de cette légèreté. C'est le cas avec le programme 380, « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires Sur la forme, nous assistons à un habituel recyclage de crédits d'un programme à un autre, d'une action à une autre. Les plus bienveillants y verront sans doute une contribution involontaire ou ironique à l'économie circulaire chère à Brune Poirson, qui, depuis lors, s'est perdue dans les limbes ... Notre rapporteur spécial Christine de nombreuses politiques menées dans le cadre du programme 380 sont des continuations des dispositifs du programme 362, « Écologie », de la mission « Plan de relance ». Concrètement, le fonds Friches est directement tiré du plan de relance, tout comme les crédits consacrés à la rénovation thermique des bâtiments, aux politiques de soutien au tri à la source et à la valorisation des biodéchets, à la prévention des risques et à l'appui aux politiques de la biodiversité. Christine Lavarde l'a parfaitement dit : la répartition des crédits au sein des trois actions du programme n'est pas détaillée dans les documents budgétaires et le financement de nombreuses politiques de fond a été détaillé après coup, soit dans la presse, soit en audition devant le Parlement. Il est tout de même incroyable que le principe de sincérité budgétaire qui, me semble-t-il, implique l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des informations financières fournies par l'État soit une fois de plus ignoré

particulièrement depuis un an, vient alimenter un flot grandissant de demandes sur la plateforme MaPrimeRénov'. Néanmoins, ce dispositif d'aide publique est grippé. Il s'apparente parfois à une boîte noire

Impossibilité de créer un compte ou un dossier, de déposer en ligne des pièces justificatives, de modifier les éléments du dossier, voilà bien des freins très concrets, qui conduisent parfois les usagers les plus précaires à renoncer. Près de

élargir l'aide, initialement réservée aux propriétaires occupants aux revenus modestes, à l'ensemble des propriétaires occupants ou des copropriétaires, puis aux propriétaires bailleurs. de grâce, il ne sert à rien d'afficher des crédits budgétaires si l'on n'est pas capable d'améliorer fortement, et surtout rapidement, la capacité opérationnelle du dispositif en fluidifiant le traitement des demandes ! Cela serait totalement contre-productif et cela viendrait affaiblir un peu plus, si si besoin était, la parole publique. Il est temps, monsieur le ministre, de mettre un peu d'ordre dans les politiques publiques. Malheureusement, il est à craindre que nous ne devions reporter nos espoirs sur le prochain PLF.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est à l'aune des retards et des manquements graves- condamnés pour certains d'entre eux -que les moyens budgétaires qui nous sont proposés doivent être appréciés. Marquent-ils, avec le passé, une rupture de l'action gouvernementale à la hauteur de la profondeur des transitions à mener ? Visiblement non, quand on constate, au terme d'une année 2022 sans précédent du point de vue des dérèglements climatiques, que ce budget est en réalité la reconduction du précédent.

2 %. Tout cela n'est pas, et de loin, à la hauteur des enjeux et de l'urgence climato-environnementale. Dans le cadre du programme 113, « Paysages, eau et biodiversité », je redis que le Varenne de l'eau est inabouti

De façon plus générale, nous devons revenir au principe de l'eau qui va à l'eau. Il est temps de supprimer le plafond mordant et d'affecter les 2,8 milliards d'euros de redevance prélevés aux agences de l'eau pour aider les collectivités et leurs syndicats à améliorer rapidement le rendement des réseaux,

Je regrette que, en première partie du budget, vous ayez refusé de donner aux communes les moyens de travailler sur les dents creuses ou sur la continuité de l'habitat des rues des villages. Il y a là, vous le savez, un potentiel d'accueil de nouveaux habitants.

vous mettez en oeuvre un bouclier tarifaire de 45 milliards d'euros, qui coûtera, net des reversements provenant des énergies renouvelables, 20 milliards d'euros. Les dispositifs sont complexes insuffisants pour les Français en difficulté, tandis que les règles d'éligibilité ont des effets de bord qui mettent en situation intenable des maires et des présidents d'intercommunalités, par ailleurs rigoureux dans leur gestion. Vous devez amplifier le chèque énergie et faciliter le retour des collectivités aux tarifs réglementés, notamment en augmentant la puissance des contrats, qui sont aujourd'hui plafonnés à 36 La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables doit aussi s'inscrire dans une planification écologique globale, dont il nous faut pouvoir, en tant que parlementaires, évaluer concrètement la cohérence et l'efficacité de mise en oeuvre. Enfin, nous sommes très inquiets des effets de l'envolée des prix de l'énergie sur la compétitivité de nos filières industrielles. On voit bien que le Président de la République peine à se faire entendre par les États-Unis d'Amérique sur la question du protectionnisme commercial. Quelles sont, monsieur le ministre, vos propositions pour restructurer le marché européen de l'électricité, dont nous voyons aujourd'hui les limites ? La parole

ce mercredi, Météo-France annonçait que l'année 2022 était la plus chaude jamais mesurée en France. Autrement dit, le changement climatique n'est pas à venir, il est déjà en cours.

le Gouvernement se trouve devant une équation quasi insoluble : il doit mener la transition écologique tambour battant, sans compromettre des finances fragilisées par un endettement record, tout en s'assurant de ne laisser personne sur le bord de la route. De fait, en caricaturant un peu, ces crédits retranscrivent une conciliation acrobatique entre le besoin d'éviter la fin du monde, tout en permettant à nos concitoyens de vivre ou, pour les plus précaires d'entre eux, de survivre, jusqu'à la fin du mois. Il ne s'agit pas de remettre en cause le bouclier tarifaire ou l'amortisseur électricité. Ces mesures sont nécessaires, en ce qu'elles permettent à nos ménages, nos entreprises et nos collectivités de lutter comme ils le peuvent contre une hausse effrénée des prix de l'énergie. Néanmoins, au vu du coût vertigineux de ces dispositifs, il faut se féliciter que les compensations habituellement versées par l'État aux producteurs d'énergies renouvelables se soient muées en recettes exceptionnelles, permettant ainsi d'en financer la plus grande partie. Cela illustre l'intérêt

Il a nécessité en 2022 l'ouverture de nouveaux crédits, pour un coût total de près de 2,9 milliards d'euros. En comparaison, 795 millions d'euros sont prévus en crédits de paiement pour 2023.

toutefois, sur son efficacité. En effet, d'après un rapport de la Cour des comptes de mars 2022, seuls 2 100 logements sont sortis en 2021 du statut de « passoire thermique », pour un objectif de 80 000. Il m'apparaît par conséquent impératif d'augmenter le taux de rénovations globales, bien plus performantes d'un point de vue énergétique que les rénovations monogestes, afin que MaPrimeRénov'soit à la hauteur des ambitions qui lui sont assignées. Enfin, je tiens à saluer vos efforts, monsieur le ministre, pour stabiliser les effectifs de votre ministère et des agences placées sous votre autorité.

les 22 milliards d'euros de crédits de paiement qui sont demandés au titre de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » en 2023 montrent à quel point l'écologie est devenue le référentiel majeur des politiques publiques. Des transports aériens, ferroviaires, fluviaux et maritimes à la reprise de plusieurs dispositifs du plan de relance, en passant par la politique de l'eau et de la biodiversité, le champ d'action de cette mission est d'ailleurs si vaste que le rattachement à l'écologie de certains secteurs interpelle. Toute politique publique a-t-elle vocation à être renouvelable, à être « en transition » et enfin à être évaluée au regard de sa performance énergétique ? Ces objectifs peuvent-ils être simplement dupliqués uniformément sur tous les territoires ? Rurales, urbaines, périurbaines, denses ou très peu denses, les communes n'ont-elles pas des spécificités qui expliquent que les modes de vie et les préoccupations de leurs habitants diffèrent ? Je me permets ces interrogations, tant il me semble que ce budget révèle une conception de l'écologie trop souvent dogmatique et étatiste. Loin du pragmatisme et du bon sens nécessaires pour répondre aux difficultés locales et les plus éloignées des métropoles, le budget de cette mission comporte plusieurs lacunes, que les rapporteurs, dont je salue le travail, ont déjà soulignées.

Les conséquences des choix du Gouvernement sur les mobilités durables sont aussi négatives quand écologie et industrie ne sont pas conciliées. Les effets pervers de la stratégie gouvernementale en matière de transition écologique du secteur automobile continuent d'apparaître. Vous me permettrez, madame Pannier-Runacher, de citer l'abandon du moteur thermique, qui a déjà produit des conséquences désastreuses sur les bassins d'emploi de l'automobile diesel, avec, par exemple, la fermeture de l'usine Bosch à Onet-le-Château, en Aveyron.

Sur ce point, il est essentiel que le Gouvernement tienne compte des modifications proposées par Christine Lavarde en tant que rapporteur spécial. Les conséquences des choix du Gouvernement sont aussi négatives lorsque le traitement de la mobilité ne tient pas suffisamment compte de la diversité des territoires. La population est de plus en plus mobile, et l'on observe des migrations pendulaires souvent contraintes, en particulier dans les territoires ruraux. L'attractivité des territoires ne se décrète pas, et le désenclavement des territoires ruraux ne peut se faire selon les méthodes qui sont appliquées dans les métropoles.

Alors que nous assistons à l'attrition du réseau aérien français, il est indispensable de renforcer le financement des aéroports de province, classés « liaisons d'aménagement du territoire ». Au total, le Grand Soir écologique dans lequel le Gouvernement veut apparaître ne trompe personne. Au contraire, il inquiète, par un dogmatisme qui peut être aveugle à la complexité des fractures territoriales. Si j'osais, je demanderais qui décide.

est votre nouveau référentiel, madame, messieurs les ministres, les solutions, même écologiques, sont plus complexes que des slogans de communication. Très bien

mois -, sa réalité, son actualité et la nécessité d'une transition vers une économie neutre en carbone et sobre dans l'usage de nos ressources naturelles. C'est plus que jamais une priorité, même si, manifestement, nous pouvons avoir

Les budgets qui vous sont présentés agglomèrent ceux du ministère de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la transition énergétique. Ils atteignent le niveau inédit de 69 milliards d'euros pour l'année 2023,

alloués à la transition écologique et 28 milliards d'euros à la transition énergétique, avec une méthode, « France Nation verte », et une déclinaison, la planification écologique, qui a fait l'objet de 22 chantiers thématiques et de 7 chantiers transversaux.

me réjouis malgré tout du million et demi de rénovations rendues possibles et des économies d'énergie et d'émissions d'ores et déjà atteintes, qui représentent l'équivalent de la consommation de la ville de Lyon.

avec une priorité assumée pour le système ferroviaire. Ainsi, plus de 6,3 milliards d'euros lui sont consacrés, soit plus de la moitié des dépenses globales en faveur des transports. Dans ce cadre, un peu moins de 100 millions d'euros sont prévus pour continuer à soutenir le fret ferroviaire.

de présenter un plan massif d'investissements dans le ferroviaire. Plusieurs dizaines de milliards d'euros sont nécessaires pour la planification écologique,

Je ne m'étendrai pas sur le secteur routier, sauf pour souligner que les budgets sont bien au rendez-vous et sont même légèrement supérieurs à la trajectoire prévue par la LOM. que la question du transport aérien, qui n'est pas taboue, reste très importante en matière d'accessibilité pour les territoires. Je veux souligner les dossiers importants qui ont progressé grâce au travail parlementaire : insonorisation des aéroports, cher Vincent Capo-Canellas, développement des lignes à grande vitesse, chers Claude Raynal, Philippe Tabarot et Henri Cabanel, ou encore taxation des carburants des jets privés, grâce au rapporteur général de l'Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, et à Jean-Marc Zulesi.

en moyenne, mais que ces taux montent parfois jusqu'à 70 %, se réjouir que le mètre cube soit bon marché ne doit pas conduire à demander à l'État de compenser les efforts qui auraient dû être faits pour assurer les interconnexions de réseaux ou la sécurisation des différents dispositifs.

C'est donc bien une progression des effectifs à périmètre constant qui vous est proposée et qui nous permettra de disposer des moyens humains de conduire cette bataille indispensable de la transition écologique. Nous allons procéder à l'examen

Tout d'abord, 2 milliards d'euros permettent de financer l'extension du périmètre du bouclier tarifaire gaz au titre de l'exercice 2022, afin de prendre en compte les structures collectives d'habitat non encore retenues par le décret du 9 avril 2022. C'est l'un

également l'extension, par un décret en cours d'élaboration, du bouclier tarifaire électricité à l'ensemble de l'habitat collectif pour le chauffage des parties communes. Les crédits ouverts doivent couvrir le second semestre 2022, ainsi que l'année 2023. À hauteur de 3 milliards d'euros, cet amendement vise à prendre en compte les moindres reversements attendus sur les contrats de soutien aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, du fait de ruptures anticipées de contrat, sur l'initiative des producteurs, qui sont intervenues depuis l'été 2022. Le Gouvernement se fonde ici sur les dernières prévisions de la CRE, parues le 3 novembre dernier, soit après le dépôt du projet de loi de finances. Ces ruptures de contrats rendront néanmoins ces producteurs redevables de la contribution sur la rente inframarginale,

Europe, fournisseurs d'énergie, nécessité de trouver des solutions ... Néanmoins, vous êtes ici dans l'une des deux enceintes du Parlement,

comme étant à même d'avoir un réel effet sur les enjeux que France Stratégie a encore soulignés. Si nous voulons atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, à savoir baisser les émissions du secteur de 50

ne lui porte le coup de grâce. Pour nous, l'adoption de cet amendement doit adresser un signal à l'ensemble de la filière et des partenaires concernés- collectivités, professionnels, locataires, bailleurs, copropriétaires -, pour leur dire que le temps est venu de réellement s'engager sur cette isolation thermique, indispensable pour la planète,

proposition se fonde sur une étude publiée en 2020 par l'initiative « Rénovons ! », qui estimait qu'un tel montant d'investissements serait nécessaire chaque année jusqu'en 2040, pour permettre au minimum la rénovation des passoires énergétiques au niveau BBC (bâtiment basse consommation)

de 2 500 logements, alors que l'on visait, il faut le rappeler, la rénovation de 80 000 passoires thermiques. Quel est l'avis de la commission ? Tous ces amendements

Une étude d'impact produite en 2020 par l'association Label Vie montre qu'un bonus au service de l'amélioration de la qualité d'accueil, du bien-être des résidents et de la protection de l'environnement permettrait aux lieux de vie engagés dans une démarche de développement durable de réduire, en moyenne, de 25 % leur consommation d'eau et de jusqu'à 70 % leur consommation d'électricité.

ainsi de financer un bonus de 1 000 euros par an pour les assistantes maternelles, de 5 000 euros par an pour les crèches et centres de loisirs et de 10 000 à 20 000 euros pour les Ehpad. Quel est l'avis de la commission

Or, ces vingt dernières années, des centaines de gares de fret et d'embranchements ferrés ont été fermés, et le nombre de cheminots travaillant à Fret SNCF est passé de 12 000 à 4 000. Afin d'enrayer cette dynamique et se fixer un objectif de 30 % du transport de marchandises transitant par le fret ferroviaire avant 2030, il convient d'investir massivement dans la relance de ce secteur, notamment au travers de la régénération et du développement du réseau d'infrastructures. L'amendement

petites lignes ferroviaires. Ces lignes du quotidien, si importantes dans nos territoires, notamment ruraux, sont depuis de nombreuses années délaissées. Pourtant, elles garantissent l'attractivité économique et touristique, ainsi

Seuls le maintien des petites lignes ferroviaires existantes, le développement d'une offre nouvelle et renforcée autour des heures de pointe dans les zones urbaines et une politique tarifaire attractive sont susceptibles d'offrir une solution de substitution crédible et effective à nos concitoyens.

à créer le débat et à répondre enfin au renouveau ferroviaire. Aujourd'hui, je défends cet amendement de la commission, qui vise à allouer 150 millions d'euros à la régénération du réseau ferroviaire. Le nouveau contrat de performance entre SNCF Réseau et l'État prévoit de maintenir un effort de régénération annuel

indispensable d'aller un peu plus loin. Tel est l'objet du présent amendement qui, compte tenu des contraintes pesant sur les finances publiques, vise à allouer 150 millions d'euros supplémentaires à la régénération du réseau ferroviaire. Comme on dit, c'est loin de faire la maille, mais cela enclenche un cycle d'investissement plus vertueux et plus ambitieux

les régions qui ne l'ont pas encore fait à rejoindre cette démarche. Nous y sommes ouverts et nous prévoirons les financements nécessaires, avec toutes celles qui s'engagent dans cette démarche dans le cadre des prochains CPER et de leur volet mobilité. D'ores et déjà, sur l'ambition de 9 000 kilomètres, plus de 6 000 kilomètres de lignes font l'objet de ces protocoles. En 2022, quelque 200 millions d'euros sont

pour avis. Monsieur le ministre, vous ne pouvez démultiplier les déclarations et les communications sur « la colonne vertébrale du ferroviaire » sans ajouter les moyens nécessaires.

Monsieur le rapporteur

monsieur le ministre,

il y a quelques jours au ministère des transports la DGITM et les différentes organisations professionnelles. Nous ferons un point au cours du premier trimestre 2023, mais je ne sais pas vous dire

voyageurs par an, dont 3,5 millions pour les lignes intérieures. Pour cela, un parc de 600 voitures de trains de nuit doit être constitué. Or le ministère des transports s'est engagé pour la construction de 300 voitures de nuit pour 800 millions d'euros. L'âge du matériel dépasse les quarante ans et la construction prend cinq ans environ. Il convient donc de financer la commande sans ajouter encore des délais supplémentaires. Cet investissement permettrait de structurer en France une nouvelle filière industrielle de construction de matériel roulant. Cet amendement, déposé par ma tend à créer un fonds d'investissement visant à reconstituer le parc de matériel roulant des trains de nuit doté de 160 millions d'euros pour sa première année. De toute évidence, nous souhaiterions qu'un montant identique soit inscrit pendant cinq ans en loi de finances, pour atteindre au total 800 millions d'euros.

pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit, et pour déployer à horizon de 2030 un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l'Europe. En 1980, la France bénéficiait d'un réseau complet, avec pas moins de 550 gares desservies par un train de nuit. À l'heure de l'urgence climatique, ce réseau constituerait un atout formidable. Un pays comme la France devrait disposer de solutions de rechange à l'avion ou à la voiture, au lieu d'accuser un lourd retard par rapport à ses partenaires européens, comme l'Autriche, qui a créé une compagnie autrichienne de trains de nuit. Ces lignes connaissent un franc succès et permettent un maillage territorial en Europe centrale et orientale qui fait largement défaut à la France.

Si nous partageons la nécessité de promouvoir et développer le transport combiné pour assurer la transition écologique, l'aide au transport combiné, dite « aide à la pince », a d'ores et déjà été réévaluée depuis 2021 de 27 millions d'euros Le montant unitaire par unité de transport intermodal versé aux opérateurs représente 31,50 euros, soit un accompagnement d'environ 70 % du coût moyen de transbordement.

925 euros pour un ménage en précarité énergétique. L'Observatoire national de la précarité énergétique préconisait en 2018 une revalorisation du chèque énergie à 710 euros,

afin de faire face à l'augmentation des factures énergétiques des ménages qui utilisent du fioul, ce qui exclut de fait les ménages ayant recours aux autres énergies hors tarif réglementé. Or les ménages résidant dans les zones rurales ont majoritairement recours à ces énergies et ne sont pas protégés

par un chauffage collectif. Cette situation est préoccupante ! Aussi, pour permettre à tous les résidents qui seraient éligibles à ce chèque d'y prétendre et de pouvoir l'utiliser, il est proposé d'abonder de 100 millions d'euros les crédits du nouveau programme ainsi créé et intitulé « Aide exceptionnelle en faveur des ménages résidant dans un immeuble équipé d'un chauffage collectif pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie ». Quel est

monsieur le ministre.

300 euros la tonne à environ 600 euros en moins d'un an. Cet amendement vise donc à créer une mesure exceptionnelle de soutien à l'achat de pellets et de bûches de bois. La dernière loi de finances rectificative a permis d'apporter une aide aux ménages touchés par cette augmentation, à hauteur de 230 millions d'euros. En se fondant sur le cours actuel des pellets de bois, nous proposons une aide à hauteur de 768 millions d'euros, qui pourra diminuer en fonction de l'évolution de l'inflation, laquelle montre aujourd'hui des signes de ralentissement.

monsieur le ministre.

par l'extension de ses missions, avec des moyens toujours plus contraints. À titre d'illustration, le projet de loi de finances pour 2023 prévoyait de diminuer de 15 millions d'euros les ressources fiscales pour le réseau des CMA et inscrivait cette baisse dans une trajectoire baissière de 60 millions d'euros d'ici à 2027, alors même que la situation de crise que nous connaissons depuis maintenant plusieurs années et le climat anxiogène qui touche nos entrepreneurs et artisans nous invitent au contraire à protéger les missions de service public de proximité des CMA. C'est pourquoi, dans la suite des amendements qui ont été adoptés en première partie, nous souhaitons que le réseau consulaire puisse bénéficier explicitement du dispositif de l'amortisseur électricité qui est prévu dans ce projet de loi de finances.

en faveur des projets de production de biogaz à partir de technologies innovantes. Un décret du 1 octobre 2021 a précisé les modalités de la procédure des appels à projets prévus dans le cadre de ce mécanisme.

du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, et dues aux anciens mineurs et à leurs ayants droit ayant souscrit un contrat de capitalisation. Il s'agit de remédier à une situation particulièrement pénalisante pour les anciens mineurs qui ont opté pour le rachat des indemnités de logement ou de chauffage dans le cadre d'un contrat de capitalisation. Au terme de l'amortissement du capital réel perçu par ces anciens mineurs dans le cadre du contrat de capitalisation, le versement des indemnités prévues aux articles 22 et 23 du décret précité aurait dû reprendre, ce qui n'a pas été le cas. Cet amendement vise donc à permettre le versement des prestations de logement et de chauffage dues et, le cas échéant, le rattrapage des montants non perçus aux anciens mineurs et à leurs ayants droit qui auraient dû en bénéficier.

Sur ce point précis, l'ANGDM nous confirme l'absence de besoin de ligne budgétaire spécifique, puisqu'un contentieux est en cours. En augmentant les crédits de l'Agence, on préjugerait de la décision de justice qui pourrait être rendue à la suite de ce contentieux intenté par certains mineurs, qui considèrent que la capitalisation n'aurait pas dû avoir comme effet de les priver de ces avantages en nature.

au régime de soutien spécifique à l'agrivoltaïsme, instauré par l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production des énergies renouvelables, qui est en cours de discussion au Parlement. de prévoir un soutien de 100 000 euros pour 2023. Ce montant est évidemment symbolique, puisque les énergies renouvelables sont actuellement davantage source de recettes que de dépenses. Les établissements visés exercent en effet des missions essentielles de formation aux réalités de l'exercice du métier d'agriculteur et aux évolutions de celui-ci. La mise en place d'installations agrivoltaïques sur leurs exploitations agricoles peut pleinement participer à ces missions.

les crédits pour soutenir la transition du parc que de les décaler dans le temps, pour qu'ils viennent en soutien de notre filière automobile lorsque celle-ci sera prête.

tendance à accepter des produits sans nécessairement demander la réciprocité. Je suis pleinement convaincu que nous devons flécher l'argent des Français vers les véhicules produits en Europe.

le coût d'une garantie de l'État à hauteur de 75 % s'élève à 150 millions d'euros. Au regard du faible taux de sinistralité observé sur le microcrédit-mobilité- environ 10 % -, un tel dispositif aurait un faible coût final pour les finances publiques : 15 millions d'euros pour ces 50 000 PTZ-m. Il s'agit donc plus d'une immobilisation de trésorerie que d'une véritable dépense

Un tel dispositif permettrait d'alléger le coût de l'achat d'un véhicule propre ou de la transformation d'un véhicule thermique et de simplifier les démarches avec une avance des aides existantes. Quel

de crédits spécifiques. Les collectivités territoriales se voient confier de plus en plus de missions sur la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine. Elles sont un acteur clé de la mise en oeuvre de la loi Climat et résilience et de la relance, les contrats de relance et de transition écologique. Sans moyens suffisants, tant en investissement qu'en fonctionnement, ces plans ne pourront pas être mis en Cette situation difficile est accentuée par la crise sanitaire et économique, qui engendre des pertes de recettes significatives pour les collectivités. Or aucun mécanisme ne permet à ce jour de savoir si les moyens de fonctionnement et d'investissement sont suffisants et efficients pour mettre en oeuvre les politiques publiques. C'est pourquoi il est proposé une enveloppe de 500 millions d'euros pour sécuriser le financement de ces contrats.

pour un total de 500 millions d'euros, le niveau de consommation des crédits semble indiquer que les crédits affectés au deuxième plan Vélo seront insuffisants pour couvrir le développement de ces usages. Avec 250 millions d'euros, il ne pourra pas atteindre l'objectif de 9 % de part modale en 2024 et de 12 % en 2030.

à l'occasion du premier comité interministériel sur le vélo, que la Première ministre présidera en début d'année, que nous déterminerons une trajectoire. Cela dit, avec 250 millions d'euros, on a largement de quoi largement investir en 2023, tant